de l'extension du domaine de la lutte- des luttes sanitaires aux combats idéologiques et politiques plus globaux. La Martinique et la Guyane sont assises au bord d'un volcan. La Polynésie française a lancé son premier préavis de grève générale. Il suffit d'une étincelle pour déclencher un brasier en Nouvelle-Calédonie, à quelques jours du référendum. L'année 2009 est toujours là pour nous instruire. Pourtant, j'estime que vous auriez pu mieux protéger Pointe-à-Pitre, livrée à elle-même. À notre demande, le Premier ministre nous a longuement reçus. Au-delà du nécessaire volet sécuritaire, pourriez-vous, monsieur le ministre, informer la représentation nationale des suites concrètes du plan d'action global, systémique et structurel annoncé, ainsi que de son calendrier à court et à moyen terme ? Face aux résistances, comment prévenir une cinquième vague et sauver des vies ? Nos collègues Bernard Jomier, Roger Karoutchi et Jean-Michel Arnaud vous ont ici fait des propositions qui pourraient vous inspirer.

cela ne va pas, nous le disons, mais, quand cela va, il faut le dire aussi ! Hier, avec le ministre des solidarités et de la santé et le secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail, vous avez présenté votre feuille de route consacrée à la prévention du mal-être et à l'accompagnement des agriculteurs en difficulté, avec un budget en hausse de 12 millions d'euros.

Monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à notre demande d'étude sur le nombre réel de suicides chaque année. C'est essentiel pour comprendre les typologies du mal-être. Ce plan progressera-t-il en reprenant d'autres propositions de notre rapport d'information ? Une évaluation des résultats est-elle prévue dans le temps ?

les mesures que nous avons annoncées hier pour lutter contre les situations de détresse agricole continueront évidemment à évoluer dans le temps. C'est bien normal et c'est ce dont nous sommes convenus. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier à mon tour, non seulement vous, monsieur le sénateur, mais également Mme Françoise Férat,

ramener les femmes à un statut d'objet, nier leur capacité à occuper leur place dans la société et, progressivement, en faisant de leur vie professionnelle et politique un enfer, les détourner des sphères de pouvoir. la clé de voûte de ce système, celle qui pourrit notre société et l'empêche d'avancer, c'est l'impunité. Celle-ci envoie aux agresseurs un message très clair, « il ne se passera rien, continuez », et aux victimes un message tout aussi clair, « on ne vous croit pas et, si l'on vous croit, on s'en fout

les actions qui tournent autour de la libération de la parole des femmes dans notre pays, que ce soit dans la sphère publique ou dans la sphère privée. J'ai lu vos doléances et j'ai surtout votre négation de toutes les actions que ce gouvernement a mises en place pour lutter contre les violences faites aux femmes depuis 2017. On peut nous reprocher beaucoup, mais ce qui est certain, et je le dis de manière factuelle et concrète, c'est qu'aucun gouvernement

C'est ce gouvernement qui a organisé le Grenelle des violences conjugales. C'est ce gouvernement qui a augmenté de 60 % le nombre de places d'hébergement pour accueillir les victimes. C'est encore ce gouvernement qui a formé plus de 90 000 policiers et gendarmes pour

les Britanniques voulaient faire le Brexit. Ils nous l'ont imposé. Nous l'avons négocié. Ils l'ont accepté. Ils veulent maintenant le renégocier. Le Brexit ne peut pas être éternel et les Européens ne peuvent pas le subir indéfiniment Après avoir tourné le dos à l'Europe, il est temps que les Britanniques assument leur choix, qu'ils assument que les trois quarts de leurs exportations de pêche dépendent du marché européen, qu'ils assument de mettre en péril une relation d'amitié, politique et économique pour 0,1 % de leur produit intérieur brut Monsieur le secrétaire d'État, il nous faut clore ce bras de fer en faisant respecter l'accord post-Brexit sur la pêche, afin que nos pêcheurs ne soient pas sacrifiés sur l'autel du Brexit. Nous demandons un engagement fort de la part de la Commission européenne. Les Britanniques jouent avec mauvaise foi sur les justificatifs prévus par l'accord de retrait.

le président Macron a décidé de les suspendre dans un souci de désescalade, pour laisser un dernier délai aux Britanniques. Le Premier ministre Boris Johnson n'a pas saisi Le Gouvernement a promis une décision avant Noël, mais le temps presse. L'annonce d'un plan de sortie de flotte sonne comme un renoncement aux oreilles des pêcheurs. Qu'en est-il de l'état d'avancement des négociations pour la délivrance des licences de pêche manquantes ? Concrètement, quelles sanctions dites croisées envisagez-vous de prendre en cas de non-réponse ? Près de deux cents de nos bateaux dépendent de l'accès aux eaux britanniques. Dans les Hauts-de-France, cet accès est encore plus important, puisque 60 % des captures de pêche proviennent de ces eaux. Il convient donc de s'assurer que les Britanniques respectent l'accord

etc. Pour construire une relation forte, même après le Brexit, nous avons besoin de confiance, nous avons besoin de lever tout malentendu, nous avons besoin de respecter les accords signés et les paroles données. C'est ce que nous faisons. Nous attendons qu'il en soit de même

parfois difficile. Le Président de la République a été extrêmement clair, nous l'avons été la semaine dernière : nous continuons ce dialogue encore quelques jours, en lui donnant sa chance, car ce serait une meilleure issue pour tout le monde, y compris pour les Britanniques, que de parvenir à une solution apaisée et concertée. Si tel n'était pas le cas, nous défendrions nos intérêts. Nous n'avons jamais hésité à le faire et à le dire et nous mettrons

la semaine dernière, la Cour des comptes a publié un rapport de vingt-deux pages qui souligne que les difficultés de notre police nationale proviennent pour l'essentiel de la mauvaise gestion des ressources humaines du ministère.

comptes constate également que les budgets de fonctionnement et d'investissement ont été fortement touchés par cette forte augmentation de la masse salariale.

ou de quelle latitude disposez-vous dans les mois qui restent avant la fin de ce quinquennat pour entamer enfin les réformes structurelles que notre police nationale attend depuis longtemps

Il a fallu six ans pour corriger cette erreur, consommatrice de crédits, moyennant quoi, il n'y avait plus de moyens de fonctionnement. Les réformes de structure, on les attend

C'est un soulagement pour les 300 employés du site, mais ne nous leurrons pas : les raisons qui ont amené le groupe allemand à envisager la délocalisation n'en ont pour autant pas disparu. En effet, le site valenciennois d'Ascoval est, comme tant d'autres, étranglé par la hausse brutale des prix de l'électricité, multipliés par trois depuis le début de l'année. Ayant choisi l'électrification plutôt que les hauts-fourneaux, ayant fait l'effort d'investir dans l'industrie verte, il en paye le prix ! Monsieur le ministre, comment expliquer à nos industriels qui jouent le jeu et s'engagent dans la décarbonation que cela se fait au détriment de leur compétitivité ? Comment justifier une telle schizophrénie de la réglementation européenne, alors même que notre mix énergétique national est parmi les plus décarbonés d'Europe ? Nous n'en récoltons pas les fruits. Au contraire, nos entreprises en sont punies Votre réponse, exclusivement budgétaire, me semble timide, ponctuelle et sans stratégie de long terme. Ascoval, comme bien d'autres entreprises, attend plus ! Permettez-moi, monsieur le ministre, de vous interroger. À l'approche de la présidence française de l'Union européenne, quelles sont les convictions que vous comptez défendre pour protéger notre souveraineté industrielle ? Enfin, quel est votre plan pour inscrire ce sujet à l'agenda et faire bouger concrètement et rapidement les choses ? À défaut, combien de délocalisations énergétiques d'ici à 2025 devrons-nous supporter ?

pour anticiper l'augmentation des coûts. La première décision, la première bataille que nous avons commencé à livrer et que je livre personnellement au Conseil des ministres européens de l'économie, c'est de découpler le prix d'électricité du prix du gaz. La France n'a pas à payer l'augmentation des prix du gaz par une augmentation de ses prix de l'électricité, alors qu'elle a des centrales nucléaires qui lui permettent d'avoir des coûts faibles de production électrique. Cela fait vingt ans qu'on le dit ! Je me battrai pour ce découplage, parce qu'il est indispensable pour l'économie et indispensable pour l'environnement. Le deuxième point, c'est de faire payer le CO2. C'est le projet, pour lequel nous nous battons, avec le soutien du Président de la République. La troisième condition stratégique, c'est de mettre en place une taxe carbone aux frontières, car nous voulons faire payer l'acier carboné à tous ceux qui veulent faire entrer de l'acier sur le territoire européen.

La compétition économique d'aujourd'hui ne se joue pas qu'avec la Chine et le Brésil. Au sein même de l'Union européenne, nous devons défendre notre compétitivité, vous venez de le rappeler. C'est une urgence.

quand allez-vous enfin prendre la mesure de la gravité de la situation et mettre en place un véritable plan ambitieux de lutte contre ces violences insupportables ?

monsieur le sénateur, me permettent de vous dire très clairement que nous avons pris la mesure du problème. Bien sûr, notre travail n'est pas terminé

d'unités de police spécialisées et surtout formées, un réel accompagnement des victimes, le renforcement de la prévention et la prise en charge des auteurs de telles violences, et ce dès le plus jeune âge. La France doit être au rendez-vous. À défaut, nous considérerions que, dans ce pays, la condition de millions de femmes vaut malheureusement bien moins de 1 milliard d'euros.

Ce lundi, un collectif composé d'employeurs et de syndicats du secteur social et médico-social, auxquels se sont associées leurs familles, s'est mobilisé pour alerter l'ensemble des parlementaires finistériens de tous bords sur la crise que connaît ce secteur d'activité. Ils étaient une centaine, réunis devant ma permanence à Lannilis. Je tiens ici à souligner la qualité de nos échanges, qui se sont déroulés dans un climat de respect et d'écoute mutuelle. Madame la ministre, mes douze collègues parlementaires

des sages-femmes au sein des établissements de santé. Le Gouvernement s'est engagé à ce que ce protocole appliqué à la fonction publique soit aussi transposé au secteur privé. Les sages-femmes territoriales bénéficieront donc des mesures de revalorisation de la grille indiciaire.

Cet accord prévoit que nos pêcheurs peuvent continuer de pêcher, notamment dans les eaux des îles anglo-normandes, s'ils répondent à un certain nombre de conditions, en particulier s'ils remplissent un critère Toutefois, les Britanniques refusent aujourd'hui d'attribuer un grand nombre de licences. Vous nous avez affirmé il y a peu, à grand renfort de formules chocs, que la France ne resterait pas les bras croisés face à cet oukase. Or, lors du G20 de Rome, le Président de la République a appelé, à la suite d'une rencontre avec Boris Johnson, « à une désescalade ». S'agit-il d'un désaveu s'agissant d'éventuelles mesures de rétorsion ? Cerise sur le gâteau, madame la ministre : la semaine dernière, vous avez annoncé brutalement et sans concertation au monde de la pêche, réuni à Saint-Pol-de-Léon, que le règlement de la crise nécessiterait un plan de sortie de flotte pour les navires n'ayant pas obtenu la licence à laquelle ils peuvent prétendre. Madame la ministre, nous sommes passés de « nous sommes prêts à leur couper l'électricité » à « nous sommes prêts à détruire nos navires pour les satisfaire ». Quel grand écart ! Le monde de la pêche est abasourdi, révolté, écoeuré

Madame la ministre, les pêcheurs réclament non pas de l'argent, mais le droit d'exercer leur métier. Cette décision, si elle était confirmée, serait inique et démontrerait une fois de plus notre faiblesse en Europe et votre incapacité à mobiliser nos partenaires de l'Union Madame la ministre, le Gouvernement confirme-t-il cette capitulation ou est-il prêt à se ressaisir et à défendre les intérêts de nos pêcheurs ?

La parole est à Mme Martine Filleul, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. de Brest à Dunkerque, 150 bateaux français attendent les autorisations pour poser leurs filets dans les eaux britanniques, onze mois mois après l'entrée en vigueur de l'accord relatif au Brexit. Face à la stratégie délibérée du Royaume-Uni de refuser l'octroi de ces licences, le Gouvernement, lui, navigue à vue. Il y a six semaines, madame Girardin, vous nous aviez demandé de vous laisser quinze jours pour préparer des ripostes. Après avoir menacé de diminuer l'approvisionnement en énergie outre-Manche, le Gouvernement a rétropédalé, arguant de la reprise du dialogue.

L'enlisement de la situation ne laisse rien présager de bon pour cette présidence. Surtout, il cause un préjudice économique et social énorme à une population fragilisée, qui ne peut plus attendre. La patience des hommes de la mer est à bout et leur colère est légitime. Sans solution gouvernementale, ils passent à l'action et envisagent des mesures de rétorsion visant les exportations vers le Royaume-Uni. Madame la ministre, trouvez-vous normal que ce soit aux pêcheurs de forcer le respect de l'accord conclu ? Combien de temps encore vont-ils être les otages de ce sabordage et payer le prix d'une crise qui est en réalité diplomatique ?

Madame la ministre, vous êtes favorable à l'utilisation du pronom « iel ». Vous avez déclaré que, pour vous, il n'était pas si choquant.

Votre position n'effacera pas les souffrances de certains parcours de vie. En revanche, elle va compliquer l'accès à la lecture des personnes en situation de handicap et de nos enfants, dont plus de la moitié n'ont pas un niveau de lecture correct à leur entrée en sixième, mais pour vous, ce n'est pas si choquant. Votre position, madame la ministre, relève de l'idéologie. « Pour moi, Pour moi, une idéologie, c'est mettre dans la tête de quelqu'un une idée qu'il n'aurait pas eue seul » : ce sont vos propos ! Madame la ministre, que fait-on en défendant la neutralité sexuelle et le pronom « iel » si ce n'est mettre dans la tête de nos jeunes des idées qu'ils n'auraient pas eues seuls ? En réalité, vous cédez vous cédez au wokisme et aux lobbies. Vous segmentez la société à coups de points médians alors que votre rôle, en tant que ministre de la République, est de défendre ce qui nous rassemble. Madame la ministre, l'écriture inclusive exclut,

qu'Édouard Philippe avait indiqué, il y a quelques années, qu'il était contre l'écriture inclusive, je me suis exprimée sur ce sujet. J'ai dit que l'écriture inclusive pouvait complexifier la compréhension de la langue française et qu'il ne fallait pas prendre cette direction, mais que j'étais totalement favorable à la féminisation des noms de métiers afin de cesser d'invisibiliser les femmes.

je vous le redis : non, je n'ai pas été choquée que le Petit Robert fasse son travail et fasse figurer dans un dictionnaire un terme qui est déjà utilisé dans la société.

Monsieur le ministre, « incompréhensible », « déséquilibré », « néfaste » : tels sont les mots utilisés par l'ensemble des acteurs du secteur aérien pour qualifier l'accord de libre-échange signé le 18 octobre entre l'Union européenne et le Qatar. Cet accord, entré en application avant même sa ratification par les vingt-sept États membres, prévoit une ouverture du ciel européen quasiment illimitée pour Qatar Airways, qui pourra ainsi desservir n'importe quelle ville, sans aucune restriction en termes de capacités ou de fréquences de vols. Certes, des droits ont été octroyés aux transporteurs européens en contrepartie, mais ils sont complètement déséquilibrés au regard du faible volume que représente la desserte de Doha. Pour le dire autrement, l'accord donne un accès illimité à un marché de 450 millions d'habitants à Qatar Airways, en contrepartie d'un accès au marché qatari de 3 millions d'habitants. Cerise sur le gâteau, l'accord prévoit également un accès au marché du fret pour cette compagnie moyen-orientale, qui pourra désormais effectuer des vols cargo directement entre l'Union européenne et des pays tiers.

vous mesurez la force du terme utilisé -obtenir de Qatar Airways le respect des règles de la concurrence, du droit social et de la transparence des comptes pour éviter notamment un dumping déguisé et le versement d'aides massives de la part de l'émirat. Rien n'étant juridiquement clair dans cet accord, il constitue un nouveau caillou dans la chaussure du secteur aérien. Après la crise sanitaire qui a mis à genoux à la fois l'industrie et les compagnies aériennes, dans un contexte où certains activistes de « l'avion-bashing » continuent d'irriguer les esprits, le secteur aérien n'avait vraiment pas besoin de cette nouvelle turbulence Monsieur le ministre, les professionnels du monde aéronautique sont très inquiets et vous invitent à ne pas ratifier cet accord, lequel est effectivement incompréhensible, déséquilibré et néfaste.

la France a fait partie des pays européens qui ont contribué à réviser la politique commerciale européenne pour la rendre moins naïve, plus affirmée, plus à même de protéger les entreprises et de prendre en compte les questions de développement durable. Pendant les semaines, les mois et les années à venir, nous allons assister à la mise en place d'instruments beaucoup plus forts pour protéger nos entreprises de la concurrence déloyale. L'accord signé le 18 octobre 2021 entre l'Union européenne et le Qatar est un accord global sur les services de transport aérien à moderniser les règles et les normes qui régissent les vols entre le Qatar et l'Union européenne. Il a été longuement négocié entre 2016 et 2019. Il comprend de nombreuses garanties. Les demandes des parties française, européenne et qatarie

Au-delà des clauses spécifiques, nous vérifierons que cet accord est bien respecté par les différentes parties prenantes. Dans le droit fil de ce que nous mettons en place d'une manière générale en matière de politique commerciale- ce que nous appelons, appelons, pour « bonne application des accords commerciaux » -, nous serons mobilisés pour faire en sorte que les engagements pris soient bien tenus et que les différentes garanties prévues dans l'accord soient respectées par les parties prenantes.

Monsieur le ministre, la situation de la Guadeloupe nous oblige. Nous réprouvons avec force toute forme de violence et affirmons que ce sont non pas les jeunes ou la jeunesse qui cassent, mais bien des délinquants. Nous exprimons notre fraternité à la population qui pâtit des blocages et des violences. Cette crise a des racines profondes que nous devons tous regarder en face. L'obligation vaccinale n'est qu'un révélateur et le sentiment de déconsidération partagé dans l'ensemble des outre-mer a été exacerbé par la centralisation des politiques publiques ces derniers mois. En effet, centraliser compte double outre-mer, car la distance accentue l'éloignement de la décision. Certes, les règles sanitaires doivent être les mêmes pour l'ensemble de la République, l'instance de dialogue annoncée par le Premier ministre est une première solution de souplesse pour gérer l'urgence. Oui, monsieur le ministre, la crise est permanente. Au fond, c'est la relation avec l'État qui se joue et la capacité des politiques publiques en général à répondre aux difficultés structurelles qui se sont empilées. 25 % des jeunes sont au chômage, un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. À cela s'ajoute l'indignité du manque d'eau potable. La majorité sénatoriale est attentive à la crise et regarde au-delà, comme elle l'a fait en 2009 en créant une mission commune d'information. Il faut en sortir par le haut, car on ne développe pas par à-coups. Le Sénat a fait des propositions solides en matière de différenciation outre-mer pour favoriser l'efficacité des politiques publiques et une relation mieux articulée entre les collectivités et l'État. Le Gouvernement est-il prêt à s'engager dans la voie d'un nouveau pacte de confiance avec les outre-mer français ?

la réplique. Monsieur le ministre, les collectivités territoriales connaissent leur territoire, et prendre en compte leur point de vue permet d'ajuster les décisions dans l'intérêt des populations locales.

Madame la ministre chargée de l'égalité, à la veille du 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, et en approchant de la fin du quinquennat, l'heure est au bilan. À ce jour, plus de 102 femmes ont été tuées en 2021, soit plus qu'en 2020. Selon la dernière étude de la Fondation des femmes, sur dix victimes de violences qui formalisent une demande, quatre n'ont aucune solution d'hébergement. Seulement 12 % des victimes de violences bénéficient d'une place et d'une prise en charge adaptée.

Plus de 22 000 femmes auraient besoin d'un hébergement pour sortir des violences, puis d'un logement social. Or, à la fin de 2021, seulement 7 820 places d'hébergement étaient disponibles, soit 1 500 de plus qu'en 2018. C'est mieux,

alors que seulement 35 % des femmes y vivent, et alerte sur la nécessité de prévoir des places d'hébergement d'urgence dans les zones rurales. L'éviction du conjoint violent, associée à l'ordonnance de protection et au téléphone grave danger, sont des avancées, mais ces mesures ne suffisent pas. Madame la ministre, partagez-vous ce bilan et ces évaluations ? Quelles réponses proposez-vous pour l'hébergement et le logement social qui soient à la hauteur des besoins de ces femmes et de ces enfants en danger ?

loin. Même si nous avons augmenté de 60 % le nombre de places d'hébergement depuis 2017, cela n'est malheureusement pas suffisant, parce que les efforts précédents n'ont pas été à la hauteur des attentes. Nous avons créé, depuis 2020,

leurs enfants. Entre octobre 2019 et septembre 2021, nous avons attribué plus de 20 000 logements sociaux aux femmes victimes de violences, soit une augmentation

pour aller encore plus loin. Nous avons mis en place un véritable plan pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'hébergement et le logement. Ce plan s'appuie sur deux axes. D'une part, nous allons former, dès le premier trimestre 2022,

et nous ferons en sorte que toutes les femmes qui ont besoin de fuir les foyers où elles subissent ces violences puissent trouver un lieu où elles se sentent protégées. Je vous remercie de votre question.

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. En ma qualité de président du groupe interparlementaire d'amitié France-Afrique de l'Ouest, je le constate avec beaucoup de regret : l'influence économique, politique, diplomatique ou même culturelle de notre pays ne cesse de se dégrader, au bénéfice d'autres pays qui, jusqu'à une période récente, ne se préoccupaient absolument pas de ce continent. Jusqu'à présent, cette situation nous préoccupait. Désormais, elle nous inquiète. Elle nous inquiète, car, progressivement, ce déclin de la France en Afrique semble changer de nature, pour se muer véritablement en un rejet, en particulier dans la zone d'intervention de Barkhane. Les rassemblements hostiles à notre pays se sont en effet multipliés ces derniers mois au Mali, au Niger, au Tchad ou, dernièrement, au Burkina Faso. Dans ce pays, le 20 novembre dernier, il y a quatre jours, un convoi des forces françaises

Malgré le sacrifice de nos soldats, malgré les succès opérationnels décisifs remportés par nos armées sur les groupes armés djihadistes, un sentiment anti-français d'une virulence inédite se développe, attisé par tous ceux qui espèrent bénéficier, d'une manière ou d'une autre, du déclassement de notre pays dans cette région. Dans ces conditions, je crains que, avant même d'avoir gagné la guerre, nous ne soyons confrontés au risque de perdre la paix. Une telle issue ne ferait que des perdants, africains comme européens, face à un terrorisme islamique qui ne désarme pas.

Il est donc urgent d'agir pour inverser la tendance. Monsieur le ministre, comment le Gouvernement compte-t-il s'attaquer à cette tâche, certes difficile, mais indispensable pour notre pays et pour l'Afrique ?

y mène. Je souhaite vous parler d'abord du convoi terrestre que vous avez évoqué. Ce convoi, qui ravitaille Barkhane, est effectivement bloqué au Burkina Faso depuis le 18 novembre.

Barkhane. Vous le savez, le Burkina Faso est aujourd'hui dans une situation sécuritaire très fragile. L'attaque d'Inata, le 14 novembre, a créé un véritable émoi dans la population : 53 gendarmes y ont été tués

L'Autriche a récemment interdit les Frères musulmans sur son territoire et, fin octobre, un rapport alarmiste a été publié sur leur financement. Dans le même temps, l'Union européenne, sans aucun état d'âme, a financé

comme un partenaire humanitaire pour la période 2021-2027, et lui a accordé 712 000 euros de subventions. Or, dans le même temps, l'Allemagne a engagé une procédure pour faire interdire les Frères musulmans de son territoire

Je vous rappelle tout de même que ces braves gens nous expliquent que les juifs sont les « petits-enfants des singes et des porcs », saluent le groupe terroriste Hamas comme « le mouvement le plus pur de l'histoire moderne encensent ses dirigeants et les décrivent comme de « grands hommes qui ont répondu à l'appel du divin sacré de la fraternité musulmane » ! Ce sont là des gens tout à fait recommandables ... Monsieur le ministre, quand allez-vous mettre un terme à ces financements ? Quand allez-vous interdire Islamic Relief Worldwide sur le territoire français ?

au cadre juridique européen. Depuis le Brexit, seule la branche armée du Hamas était considérée comme terroriste dans le droit britannique. La décision récente étend cette mesure à l'ensemble du mouvement, ce qui ne fait que rejoindre le droit applicable depuis longtemps dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Sur la question plus large des mouvements radicaux antisémites, appelant à la haine ou à la violence, je veux rappeler la fermeté absolue du Gouvernement. Celui-ci a pris la décision de dissoudre plusieurs associations présentes sur le territoire national,

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, l'examen en nouvelle lecture de ce second projet de loi de finances rectificative pour 2021 fait suite à l'échec de la commission mixte paritaire. mixte paritaire. Le compromis n'était pas aisé, étant donné que vous aviez supprimé, en première lecture, l'ensemble du dispositif d'indemnité inflation annoncé par le Premier ministre pour garantir le pouvoir d'achat des Français.

Je constate aussi que l'Assemblée nationale a souhaité revenir sur les dispositions fiscales introduites par le Sénat en matière de TVA au titre de la consommation d'électricité, d'éligibilité des sociétés de capital-risque au PEA-PME,

de loi de finances rectificative est un marqueur de notre sérieux budgétaire, puisqu'il contribue à financer les besoins de fin de gestion de l'État. Grâce à l'effet conjoint de la révision à la hausse de la croissance, de l'annulation des surplus de crédits d'urgence et de la maîtrise des dépenses ordinaires- celles-ci

Ce projet de loi de finances rectificative contribue à garantir la protection des Français, à favoriser la relance de l'économie, notamment à travers les redéploiements du plan de relance, et à préparer l'avenir par la mobilisation d'un certain nombre de dispositifs. Je suis heureux que ce texte puisse poursuivre son parcours parlementaire,

attendre dans le cadre d'un collectif budgétaire de fin de gestion. Malheureusement, rien n'est fait en revanche pour s'attaquer au désendettement.

et des minima sociaux visés par l'indemnité inflation, soit 3,9 millions de personnes, ce qui inclut les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité, ceux de prestations versées par l'assurance chômage, qui devaient être prises en charge par la mission « Travail et emploi » dans le dispositif proposé par le Gouvernement, et les 600 000 bénéficiaires du minimum vieillesse. En outre, les crédits ouverts à hauteur de 50 millions d'euros sur la mission « Travail et emploi » permettraient aux opérateurs de la politique de l'emploi d'attribuer, au cas par cas et en fonction des besoins, des aides en faveur des demandeurs d'emploi et des jeunes en parcours d'insertion,

Elle a par ailleurs procédé à quelques ajustements sans grande incidence aux articles 3 et 6. Les députés ont également modifié l'article 8, en adoptant un amendement du Gouvernement tendant à rehausser

L'Assemblée nationale a également conservé l'article 14, qui confirme, en l'inscrivant dans le code de l'action sociale et des familles, l'exclusion des primes liées à la performance versées par l'État aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux Paralympiques

après l'échec prévisible de la commission mixte paritaire, nous réexaminons ce deuxième projet de loi de finances rectificative en nouvelle lecture. Son issue fait peu de doute, puisque M. le rapporteur général a déposé une motion tendant à opposer la question préalable, comme il est souvent d'usage à ce stade de l'examen

La bonne nouvelle, dont il faut se réjouir, est que l'acquis de croissance en 2021 laisse d'ores et déjà augurer une fin du rattrapage économique de la crise déclenchée par la pandémie d'ici à la mi-2022, toujours si l'on en croit les prévisions. La moins bonne nouvelle, c'est que la gestion de cette crise inédite s'est faite au prix d'un creusement considérable des déficits, avec des aides souvent utiles, mais qui posent aussi parfois question, comme le soutien direct à certains secteurs économiques sans conditionnalité sociale ou environnementale. Il reste que l'État a joué son rôle d'amortisseur en temps de crise, alors que la lutte contre le coronavirus reste une priorité- plus de 30 000 nouveaux cas d'infection ont encore

de relance » pour soutenir le réemploi des déchets, ou encore ma proposition de conditionner le remboursement des prêts garantis par l'État (PGE) à la capacité réelle des entreprises à rembourser. Je salue néanmoins les renforts de personnels décidés dans certaines administrations pour faire face aux conséquences du Brexit,

En première lecture, mon groupe avait voté contre la suppression de l'article 12, considérant, bien que la mesure soit discutable, et surtout coûteuse, qu'il était désormais difficile de revenir sur une telle annonce.

pouvoir d'achat ; la compensation des pertes tarifaires des régies locales, qui affectent particulièrement ces structures et les collectivités dont elles dépendent ; enfin, le prolongement du fonds de solidarité à L'enjeu majeur de ce budget rectificatif est le déploiement du plan de relance, en particulier son tuilage efficace avec les mesures d'urgence, la consommation effective des crédits votés et la réception du volet européen de 40 milliards d'euros. ombre au tableau, la moindre lisibilité des crédits autorisés, avec des reports très importants entre 2020 et 2021. Il est vrai que nous avions voté pas moins de quatre collectifs budgétaires l'an dernier ! De tels reports seront-ils

Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour en discuter, après la réunion d'une commission mixte paritaire qui fut, sans surprise, non conclusive. La question du pouvoir d'achat est majeure en ces temps de crise. D'ailleurs, le groupe socialiste a proposé de nombreuses mesures redistributives

ministre, nous n'avons pas validé non plus le dispositif proposé par la majorité sénatoriale, car, en fait, nous avions le choix entre deux dispositifs de droite ! Le chèque inflation du Gouvernement

Son objectif principal était avant tout de faire des économies, et elle laissait de côté la question de l'accès aux droits, sans répondre durablement à l'urgence sociale. Nous avons déjà eu l'occasion de le dire dans cette enceinte : les 3,8 milliards d'euros que l'exécutif consacre au soutien du pouvoir d'achat ne nous posent aucune difficulté. Au contraire, ce montant pourrait même se révéler insuffisant pour soutenir véritablement ceux de nos concitoyens qui se trouvent en difficulté du fait des hausses du prix de l'énergie, des carburants et des denrées alimentaires. Nous refusons que nos concitoyens s'enfoncent dans la précarité. Nous souhaitons une remise à plat de la fiscalité et de la redistribution, seule à même d'assurer aux Français les plus modestes les moyens de vivre dignement dans un contexte économique difficile. Je regrette que toutes les propositions que nous avons pu faire en ce sens durant ce quinquennat aient été balayées d'un revers de la main. Pourtant, ces 3,8 milliards d'euros, que l'on trouve si dispendieux dans cet hémicycle, ne représentent pas grand-chose à côté des avantages fiscaux généreusement accordés.

La situation de plusieurs millions de personnes dans notre pays ne cesse de se dégrader. Des mesures structurelles sont à prendre d'urgence. Le dispositif gouvernemental et son alternative sénatoriale ne sont pas à la hauteur des enjeux. Mais, bien entendu, nous n'avons pas la même façon d'appréhender la justice sociale et la justice fiscale. Dont acte. Néanmoins, acte. Néanmoins, qui peut s'opposer à un coup de pouce, quelle qu'en soit la forme, quel qu'en soit le montant, singulièrement à l'approche des fêtes de fin d'année ? La réponse est évidente Maintenant, au-delà des grands discours, j'aimerais bien connaître les propositions structurelles du Gouvernement et de la majorité sénatoriale pour soutenir le pouvoir d'achat et lutter contre les inégalités. En ce qui nous concerne, cela fait des mois que nous avançons des propositions concrètes de redistribution des richesses en cette période de reprise de la croissance. Comme lors de son examen en première lecture, nous nous abstiendrons donc sur ce texte.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'échec de la commission mixte paritaire, lundi dernier, n'aura surpris personne, car les désaccords constatés étaient trop importants. Le Sénat a en effet supprimé l'indemnité inflation proposée par le Gouvernement et votée par l'Assemblée nationale, prétendant qu'il s'agissait d'une mesure électorale et qu'elle relevait du bricolage budgétaire. Mais, si c'est le cas, mes chers collègues, comprenez que je m'étonne que vous ayez choisi de la remplacer par un dispositif bricolé à la hâte avant la séance Et là, miracle de la discussion budgétaire : une fois reprise par la majorité sénatoriale, ce n'est plus une mesure électorale ni du bricolage budgétaire, mais une mesure attendue par nos concitoyens

J'ajoute que la critique d'un prétendu « chéquier de campagne » n'est pas nouvelle. Faudrait-il donc que nous renoncions à réformer et à financer les politiques publiques

pour ne voir dans la réponse de l'État qu'une mesure électoraliste ? Et quand le Président de la République avait annoncé la fameuse prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en 2018, pour répondre à la colère exprimée par nos concitoyens, était-ce déjà un cadeau de campagne ? Cela ne tient pas debout !

nous n'en discuterons pas ! L'Assemblée nationale a également retenu l'article 13, introduit par le Sénat, et a même proposé de l'enrichir pour prendre en compte, en plus des besoins spécifiques de La Réunion, la situation particulière de la Guadeloupe et de la Martinique. Mais nous n'en discuterons pas ! Elle a rétabli le financement de l'activité partielle de longue durée, dont je rappelle que votre collègue Éric Woerth avait salué l'utilité dans son rapport sur la mission « Plan de relance ». Mais nous n'en discuterons pas non plus ! Pourtant, nous sommes nombreux à avoir critiqué votre proposition de remplacer le chèque inflation. Nous avons tous déploré que votre proposition mette à l'écart les travailleurs indépendants, les retraités, les demandeurs d'emploi ou encore les étudiants boursiers. Selon vos propres chiffres, elle écarterait plus de 33 millions de Français d'un dispositif de soutien.

Vous nous dites que le Gouvernement dépense sans compter, mais nous aurons effacé en deux ans plus des deux tiers du déficit dû à la crise, quand, dans le même délai, ... Veuillez conclure. ... ceux qui étaient en responsabilité durant la crise de 2008 n'avaient fait que la moitié du chemin. Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI soutiendra le Gouvernement et le pouvoir d'achat des Français

Cette année, ce texte nous arrive après un semi-marathon, ou plutôt après un abandon à mi-parcours. À la suite de l'explosion en plein vol du projet de loi de finances pour 2022, je ne donne pas cher du présent Et pour cause, en cette période de précampagne électorale, tout texte disposant d'un contenu politique, aussi minime soit-il, fait l'objet d'un examen brouillé par les enjeux des prochaines échéances. En l'espèce, la situation est assez claire : la commission mixte paritaire a achoppé sur l'article 12 de ce budget rectificatif, qui prévoit l'instauration de l'indemnité inflation.

Au fond, la question qui nous est posée au cours de cette séquence budgétaire est la suivante : à quoi sert le Sénat ? À quoi sert le Sénat en période budgétaire ?

Sur ce sujet comme sur bien d'autres, le Sénat ne peut avoir le dernier mot contre l'Assemblée nationale. C'est dommage, mais c'est ainsi ... Partant de ce constat, comment

d'obtenir gain de cause sur certains sujets clés ? La Constitution de la V République nous assigne le second rôle et, finalement, qui n'est pas satisfait de cette situation peut parfaitement se présenter à l'Assemblée nationale du texte qui nous intéresse aujourd'hui, le Sénat a posé de bonnes questions, mais n'apporte pas les bonnes réponses. Le dispositif de l'indemnité inflation était-il bien calibré ?

du cours des carburants. Vous introduisez une discrimination entre des foyers fiscaux qui présentent pourtant des situations financières très différentes : ainsi, un couple dont l'un des membres gagne le SMIC et l'autre

Le Gouvernement et sa majorité ont eu beau jeu d'attaquer le Sénat, en répandant la fausse rumeur selon laquelle nous aurions purement et simplement refusé d'accorder à 38 millions de nos concitoyens une indemnité de 100 euros.

Si nous avons fait le choix de supprimer l'article 12, c'est pour lui préférer un dispositif mieux ciblé, plus efficace et moins coûteux. La commission des finances, par la voix de son rapporteur général, propose une mesure simple, qui s'appuie sur des outils existants

Le Gouvernement ne s'est pas complètement opposé à cette mesure : il a prévu un régime transitoire en instaurant un taux de réfaction de 35 %, qui reviendra au taux actuel de 25 % en 2024. C'est un petit pas que je tiens tout de même à saluer.

d'une mesure de bon sens que nous avons été très nombreux ici à voter. Je me réjouis qu'elle figure dans le texte adopté hier soir par nos collègues députés.

à 8,2 %. Soulignons que les dépenses ordinaires ont augmenté de 41 milliards d'euros entre 2020 et 2021, soit deux fois le montant des mesures d'urgence et de relance. Je signale également que le déficit budgétaire de l'État s'établira à 205 milliards d'euros en 2021, avec près de 24 milliards d'euros de crédits non consommés en 2020 et reportés en 2021. Je n'aurai pas l'indélicatesse de rappeler les observations sévères du Haut Conseil des finances publiques, qui regrette que le maximum n'ait pas été fait au cours de cette année pour contribuer au désendettement de notre pays. Au fond, monsieur le ministre, le texte que nous nous apprêtons à rejeter ce soir répond à la même logique que le texte que nous avons rejeté hier dans le cadre de

un endettement qui s'aggrave, année après année, menaçant d'avance la prospérité des générations futures. Enfin, nous ne pouvons accepter de voter un texte qui comporte une mesure coûteuse et démagogique, alors que nous avions proposé, ici même au Sénat, une solution de bon sens qui garantissait aux ménages modestes un soutien financier plus important et mieux ciblé. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains votera la motion présentée

Parmi elles se trouvent une grande majorité de mères célibataires, mais également des étudiants et des autoentrepreneurs, contraints de choisir entre se chauffer, se nourrir ou se soigner. Les mobilisations en Guadeloupe et à la Martinique- je parle bien des mobilisations et non des comportements qui, à mes yeux, ne sont pas des actions revendicatives -sont symptomatiques de la détresse sociale, à laquelle ce Gouvernement n'a su apporter que des réponses peu ambitieuses,

subissent des contrôles de plus en plus fréquents et déshumanisants. Cette politique pour les riches, grands gagnants de ce quinquennat, est à l'opposé de celle que nous défendons. En d'autres termes, la dignité des uns s'arrête là où commencent les dividendes des autres ... Tant sur le fond que sur la forme, ce texte et les débats budgétaires qui l'ont entouré sont loin d'être à la hauteur.

sans surprise, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du second projet de loi de finances rectificative pour 2021 n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte de compromis.

voilà encore seulement quelques semaines. Au-delà de ce rebond de croissance, il y a sans doute d'autres causes à l'inflation. Pour endiguer l'effet de surchauffe, les Français réclament des mesures tout à la fois rapides, fortes et efficaces, solutions qu'il conviendrait d'apporter sans être trop dispendieux : il va falloir résoudre la quadrature du cercle.

Ce problème subsiste dans le texte adopté par le Sénat, qui exclut toute une catégorie de revenus, compris approximativement entre 1 500 et 2 000 euros. Il exclut également des catégories entières de bénéficiaires

C'est cette raison qui avait poussé, en première lecture, le groupe Union Centriste à s'abstenir sur ce collectif budgétaire. Nous l'avons fait à regret, car nous avions jusque-là voté les différents budgets rectificatifs qui visaient à faire face aux conséquences de la crise sanitaire.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

dans la prochaine loi de programmation, au moment même où nous nous prononçons sur des projets de lois de finances comportant des mesures dispendieuses, y compris pour l'avenir. Mais je n'y reviens pas. Par-delà ces considérations d'opportunité, je veux saluer l'accord que nous avons trouvé avec nos collègues députés. Les textes comportent des améliorations notables, qui faciliteront l'examen et le contrôle des prochains budgets. Ils conservent des apports substantiels du Sénat, que nous avions notamment défendus, le président Claude Raynal et moi-même, en tant que rapporteurs lors de la première lecture. Ainsi, la fixation d'une norme pluriannuelle de dépenses des administrations publiques est une bonne chose. chose. Maîtriser la dépense publique est indispensable si l'on veut retrouver un second souffle budgétaire. Le texte que nous avons établi, fruit d'un compromis, n'a malheureusement pas retenu notre proposition d'une loi de programmation rectificative. les lois de programmation feront bien l'objet d'une présentation par catégorie d'administration publique, et comprendront trois scénarios d'évolution des taux d'intérêt, avec leurs conséquences sur la charge de la dette.

Le débat unique qui regroupera à la fois celui sur le programme de stabilité et le débat d'orientation des finances publiques est également bienvenu, dès lors que, comme le souhaitait, là encore, le Sénat, il peut se dérouler en avril, avant la transmission du programme de stabilité à la Commission européenne. nous avions considéré que ce moment « pluriannuel », consacré aux grandes orientations budgétaires, pouvait aussi être celui du débat sur la dette, que l'Assemblée nationale, pour sa part, et assez légitimement, souhaitait plutôt pour la rentrée de septembre, avant l'examen du projet de loi de finances. Une solution de compromis a permis de concilier les spécificités du travail des deux assemblées, ce dont je me réjouis.

Des dispositions ont par ailleurs été adoptées, sur notre initiative, afin de mieux encadrer l'exécution budgétaire et de renforcer le contrôle et l'information du Parlement. Ainsi en est-il de la limitation des reports de crédits,

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs,

La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) a fêté son vingtième anniversaire le 1 août dernier. Grâce à elle, et depuis près de deux décennies, le Parlement et les gouvernements successifs ont travaillé à rendre la programmation et la gestion des finances publiques plus démocratiques et plus performantes. À l'occasion de cet anniversaire, nous pouvons donc saluer les fondateurs de la LOLF, Alain Lambert et Didier Migaud, qui ont grandement contribué, par leurs travaux et leur détermination, à améliorer notre architecture budgétaire. budgétaire. Vingt ans plus tard, le bilan est sans équivoque : la LOLF est une vraie réussite. Tout d'abord, elle a approfondi à bien des égards les droits du Parlement. Pour ne citer que quelques exemples, celui-ci examine et vote les moyens de l'État par politique publique et non plus par budget des ministères. Nous discutons ainsi de la destination réelle des crédits, ce qui n'était pas le cas avant 2001, bien que cela soit essentiel pour faire la transparence sur l'usage de la contribution publique. Par ailleurs, le Parlement vote la totalité des crédits de chaque mission budgétaire, ce qui n'était pas non plus le cas avant la LOLF, car, je le rappelle, les crédits de l'année précédente étaient simplement reconduits par un vote unique. Enfin, les parlementaires peuvent amender les crédits budgétaires, ce qui constitue une amélioration notable et profonde du droit d'amendement. Il s'agit aussi d'une réussite en ce qui concerne la performance de la dépense publique. Les progrès apportés par ce texte sont indéniables à cet égard. Le Parlement dispose d'un outil précieux pour évaluer la performance, en l'occurrence la documentation budgétaire qui est, en France, l'une des plus riches au monde. Pour autant, malgré ces succès et ces avancées, la pratique n'a pas épuisé l'ensemble du potentiel de la LOLF. Nous devons nous saisir de tous les moyens qu'elle met à notre disposition. Beaucoup a été fait pour que les règles de comptabilité et de gestion budgétaires accompagnent le mouvement de la LOLF, mais nos efforts doivent se poursuivre, tant du côté du Parlement que du Gouvernement.

Le Gouvernement a contribué à la réflexion, notamment en demandant à la commission sur l'avenir des finances publiques, présidée par Jean Arthuis, de faire des propositions sur les questions de gouvernance des finances publiques. Elle a rempli sa mission, qui, je le pense, a été d'une grande utilité. Le Sénat a activement participé à ces travaux. Je salue à cet égard l'action du rapporteur général et du président de la commission des finances. Je me réjouis de l'accord conclu en commission mixte paritaire, car il traduit l'équilibre institutionnel qui a été trouvé en dépit des divergences politiques. La proposition de loi organique qui en ressort constitue une avancée majeure pour le pilotage de nos finances publiques. Elle consolide les pouvoirs du Parlement en apportant une pierre supplémentaire à l'entreprise d'amélioration de la qualité et de l'efficacité de la discussion budgétaire, au service de la maîtrise de nos finances publiques. premier objectif que vise le texte dont nous débattons est d'insérer une dimension pluriannuelle dans la discussion budgétaire. C'est un apport essentiel aux yeux du Gouvernement. Le deuxième objectif est de continuer à renforcer la sincérité des lois financières. Si la présente proposition de loi organique est adoptée, le Gouvernement devra justifier les éventuelles déviations de la trajectoire prévue

prévue l'organisation d'un débat sur la situation des finances locales, sur l'initiative du Sénat, et d'un débat sur la dette publique. Pour ce qui concerne le cadrage général, le débat d'orientation des finances publiques sera refondé. S'y substituera une obligation pour le Gouvernement de fournir au Parlement les plafonds de crédits par mission dès l'été. Ainsi y aura-t-il un débat unique portant sur l'orientation des finances publiques. Enfin, cette proposition de loi organique a été enrichie par les débats parlementaires et la commission mixte paritaire. paritaire. Par exemple, la LPFP et l'article liminaire devront comporter une prévision de dépenses d'investissement, ce qui permettra de mieux définir ces dépenses et de les identifier.

recourant à la dotation relative aux dépenses accidentelles et imprévisibles, le Gouvernement doit en informer les commissions des finances trois jours au moins avant la publication de l'arrêté ouvrant ces crédits. Nous comprenons cette exigence d'information et de transparence. Néanmoins, il faut être prudent, car cette dotation est faite pour faire face à des besoins d'urgence. Or on ne peut pas exclure qu'à l'avenir une situation d'une urgence exceptionnelle nécessite une ouverture massive et très rapide de crédits. Il s'agirait d'une urgence telle qu'il serait impossible d'attendre trois jours sans que cela ait des conséquences extrêmement néfastes. Aussi, nous pensons que, dans ce cas très restreint, une certaine souplesse devrait s'appliquer.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

modifier la LOLF, avec pour objectif affiché d'améliorer l'information du Parlement sur les finances publiques, nos outils d'analyse, et de réorganiser la discussion parlementaire de nos lois financières pour en assurer une meilleure lisibilité.

Chacun de nous étant soucieux d'améliorer le travail parlementaire, il n'était pas difficile de trouver un terrain d'entente sur un certain nombre de points, même si, sur le fond, nous trouvons, pour notre part, que les apports de ce texte restent trop limités.

avec des règles européennes qui auront peut-être évolué d'ici là. Nous nous étions d'ailleurs interrogés en septembre dernier sur la réelle nécessité d'inscrire l'examen de ces textes à l'ordre Au moins, aujourd'hui, le calendrier du Sénat n'est pas encombré ; profitons-en pour faire aboutir ce texte dont l'initiative revient, rappelons-le, à l'Assemblée nationale.

En somme, même si nous saluons la qualité des débats, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, et la volonté commune de moderniser la LOLF sans la vider de son sens ni de son esprit, organique reste une occasion partiellement manquée de rendre possible un débat collectif annuel sur l'ensemble de nos choix collectifs, c'est-à-dire aussi sur le niveau de la fiscalité, la redistribution et les grands enjeux auxquels l'État peut répondre. Les auteurs de la proposition de loi organique affirment qu'elle est « politiquement neutre » et sans impact sur la nature des choix politiques qui seront faits à l'avenir. Ce n'est pas tout à fait vrai, car la discussion budgétaire se concentre sur les dépenses et la dette, comme si les ressources de l'État ne pouvaient pas, elles aussi, être pilotées. Reconnaissons néanmoins que ce texte évite finalement des dispositions plus contraignantes et controversées, qui n'auraient pas été acceptables de

Nous saluons le travail accompli de longue date dans ce domaine. Je pense tout d'abord à la mission d'information de la commission des finances de l'Assemblée nationale sur la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances.

Il appartiendra aux pouvoirs publics de s'emparer de ce nouveau cadre organique. Comme cela a déjà été précisé, ce cadre redéfini ne s'inscrit aucunement dans une politique d'austérité, mais vise à atteindre un objectif bienvenu d'efficacité et de lisibilité. Parmi les ambitions de la LOLF figurait le passage d'une logique de moyens à une logique de résultat. Ce développement d'une culture de la performance passait par une plus grande responsabilisation des gestionnaires et par une indispensable réduction des dépenses de l'État. ans après, force est de constater que la LOLF n'a pas été un outil aussi efficace que l'on aurait pu l'espérer pour endiguer les déficits successifs et que les gestionnaires publics n'ont pas pleinement su adopter cette culture de la performance. Il nous reste encore du chemin à parcourir Il nous faudra également renforcer les liens entre l'examen du budget de l'État et le suivi des dépenses de sécurité sociale et de celles des collectivités, dont le montant cumulé dépasse de loin celles de l'État. Il nous faudra également renforcer le rôle du Parlement et les pouvoirs d'évaluation et de contrôle des deux commissions des finances, afin de rendre possible un véritable chaînage vertueux entre l'évaluation des résultats passés, l'autorisation budgétaire pour l'année à venir, la programmation pluriannuelle et l'exécution en cours d'année. Cet esprit animait, il y a vingt ans déjà, les fondateurs de la LOLF ; il devra continuer de nous animer dans les années à venir. En dotant notre constitution financière d'outils nécessaires aux pouvoirs publics, ces dispositions, une fois adoptées, permettront de gérer plus convenablement les nouveaux enjeux propres aux finances publiques, issus de la crise de la covid-19. partager les objectifs défendus, à savoir un meilleur pilotage des dépenses et de la dette publiques, organisé de façon pluriannuelle, une application plus stricte de nos principes budgétaires et un rôle accru du Parlement dans le contrôle des politiques publiques en la matière. Plusieurs compromis ont ainsi pu être trouvés, notamment sur la discussion des taxes affectées, le calendrier respectif du rapport et du débat sur la dette publique, ou encore la distinction entre investissement et financement. La recherche du compromis est toujours nécessaire. Le trouver est toujours une satisfaction. Rappelons qu'il n'est possible que lorsqu'il y a débat ! La parole est à M. Emmanuel Capus, pour le groupe Les Indépendants

d'une part, une proposition de loi organique visant à modifier la loi organique relative aux lois de finances, d'autre part, une proposition de loi ordinaire relative au Haut Conseil des finances publiques. En cette période budgétaire quelque peu houleuse, l'examen de ces deux textes fait l'effet- pour nous tous, je crois -d'un havre de paix au milieu d'une mer agitée. Tâchons d'apprécier le moment : je doute qu'il y en ait d'autres cette année ! À quelques mois de l'élection présidentielle, il n'est pas commun de faire émerger un tel consensus, qui dépasse les clivages ordinaires entre les deux chambres comme entre les groupes politiques. Je tiens à cet égard à saluer le travail sérieux et courageux mené de concert par le rapporteur général et le président de la commission des finances. Au fond, la raison de ce consensus est assez simple : ces deux textes ne fixent pas, à proprement parler, ne fixent pas, à proprement parler, de cap politique ; ils redéfinissent plutôt le cadre dans lequel ont lieu les débats sur la politique budgétaire. Pour user d'une métaphore sportive, il s'agit là de changer les règles du jeu et non de jouer un match. Sans surprise, ces débats soulèvent donc moins de passions que les textes budgétaires ordinaires, mais ils n'en sont pas moins importants. Plus fondamentalement, comme j'avais eu l'occasion de le dire en septembre dernier lors de la première lecture, je crois que ces deux textes marquent trois avancées majeures pour l'orientation de nos finances publiques. La première La première avancée, c'est un renforcement, dans les documents budgétaires, de la distinction entre dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement. Pour beaucoup d'élus locaux, cette distinction tombe sous le sens, car ils la font au quotidien dans leur collectivité. Je suis satisfait que le Parlement s'inspire de cette bonne pratique, qui est issue, si je puis dire, du terrain. La deuxième avancée, c'est une révision du calendrier budgétaire à l'aune de la pratique parlementaire. Là encore, je crois que ces textes tirent les bons enseignements de deux décennies d'examen des textes budgétaires dans le cadre fixé par la LOLF. En particulier, la suppression du débat d'orientation des finances publiques et la création d'une nouvelle catégorie de lois de finances pour clore les exercices budgétaires vont dans le bon sens ; ils n'ont d'ailleurs guère soulevé de débats. Je me réjouis aussi que notre assemblée puisse se prononcer régulièrement sur la soutenabilité de notre dette publique, ainsi que sur la situation financière des collectivités. La troisième et dernière avancée, c'est un renforcement de la programmation des finances publiques. J'espère que cette nouvelle pratique nous permettra enfin de mieux piloter nos dépenses et nos investissements sur le temps long et de résorber ainsi notre déficit public. Il s'agit en effet d'un préalable indispensable pour engager, dès le début du prochain quinquennat, la diminution de notre dette publique. Vous l'aurez compris, notre groupe votera ces deux textes, qui vont dans le bon sens. Pour conclure, mes chers collègues, je me permets de partager avec vous une remarque de fond sur le calendrier assez improbable de ces deux textes. Il est en effet saisissant que nous décidions de renforcer la programmation de nos finances publiques, alors même que nous sortons à peine d'une crise sanitaire et économique dont personne n'avait prévu l'ampleur. Autrement dit, c'est après avoir constaté que la dépense publique a quelque chose de fondamentalement imprévisible que nous choisissons de renforcer l'effort de prévisibilité. C'est bien ce que nous avons dit au Gouvernement ! Espérons que ces textes nous aideront effectivement à assainir nos finances publiques.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous avions dénoncé avec force l'introduction d'une gestion pluriannuelle des finances publiques lors de l'examen en première lecture de la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. pas par refus d'anticiper l'avenir ou par rejet d'une forme de planification des politiques publiques. En effet, les enjeux actuels, tout particulièrement les enjeux climatiques, appellent à s'extraire de la vision court-termiste d'un capitalisme productiviste qui place la recherche absolue du profit immédiat au-dessus de toute chose.

au profit d'un petit nombre de privilégiés qui n'ont cessé d'être favorisés pendant ce quinquennat. Force est de constater que la commission mixte paritaire n'a pas oeuvré à changer l'orientation de ce texte. Sans aucune considération pour la nécessité de réaliser des investissements d'avenir, consacre un autosabotage des capacités d'intervention de l'État, pourtant indispensables à la transition écologique. Alors que la nouvelle donne de l'urgence climatique aurait pu nous inviter à définir de nouveaux indicateurs de l'action publique, on persiste ici à ne concevoir la richesse de la société qu'à travers le seul PIB.

Les Français devraient pourtant avoir le droit de savoir à qui ils versent chaque année des intérêts ; il faudrait aussi prévenir toute tentative de concentration des avoirs à des fins de pression politique.

Nous ne pouvons cacher notre étonnement quant au soutien de la majorité sénatoriale à cette disposition, qui vient consacrer la supériorité d'une instance technocratique, non élue, sur le Gouvernement et le Parlement. À croire, mes chers collègues de la droite, que votre obsession commune pour la réduction des dépenses publiques prend le pas sur la démocratie parlementaire Aucune leçon ne semble avoir été tirée du fait que c'est bien la hausse des dépenses publiques qui a permis de réduire l'ampleur de la crise économique et sociale déclenchée par l'épidémie de la covid-19.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, sans surprise, c'est dans un consensus total que les rapporteurs et présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat se sont accordés sur un texte prétendant « moderniser la gouvernance des finances publiques ».

tous le rôle marginal du Parlement dans le processus budgétaire, à cause tantôt de l'article 40 de la Constitution, tantôt de la fongibilité asymétrique. Face à toutes ces préoccupations que nous avons en commun et auxquelles ce texte n'apporte aucune réponse, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste a transcrit ses conclusions dans plus d'une vingtaine de propositions.

et contribue à écarter encore davantage le Parlement des débats budgétaires. Nous tenons à exprimer notre profond désaccord sur l'instauration de la pluriannualité à des fins de réduction des dépenses publiques. Il ne s'agirait que d'un « outil », d'un « cadre

de favoriser telle ou telle orientation politique. Il ne s'agit évidemment pas d'un texte austéritaire, mais d'un nouveau cadre amélioré de nos discussions, afin que celles-ci soient les plus transparentes et les plus efficaces possible. Chaque gouvernement restera évidemment libre de mener la politique pour laquelle il aura été élu. » Comme si notre opposition au texte était due à notre incompréhension ! Mes chers collègues, nous avons bien compris ce que signifie la pluriannualité. L'introduction, dès les premiers mots de ce texte, de l'expression « dans dans le respect de l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques », objectif inscrit déjà depuis 2008 dans la Constitution, vient cadenasser les pratiques et contrevient aux décisions politiques ultérieures. Vous faites d'un débat politique et économique un choix de principe, fondé sur un postulat. Déjà présente à onze reprises- onze ! -dans la LOLF, la notion d'«

! Sous prétexte d'une dette publique érigée en problème économique fondamental, ce texte consacre le dogme libéral dans les principes budgétaires. Franck Waserman, professeur de droit public, l'explique : « L'équilibre apparaît davantage comme un paramètre économique que comme un principe structurant qui puisse se couler dans les formes du droit. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles il n'a jamais été formalisé sous forme d'un principe juridique des finances publiques, et qu'il n'a probablement pas vocation à l'être un jour. » Les indicateurs ne constituent pas des outils et leur multiplication façonne la vision des politiques, des médias et de la société.

lui-même que ce type d'indicateur constituait « un recul de la transparence démocratique ». En plus d'être inopérants et vecteurs d'une idéologie austéritaire, ces indicateurs ajoutent donc de l'illisibilité à la confusion.

L'adoption en commission mixte paritaire d'un texte de compromis sur la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques rappelle l'importance de tenir cet objectif, qui transcende les divergences politiques. Ces évolutions organiques font écho au rôle essentiel de la représentation nationale en matière de finances de l'État. Je l'ai rappelé hier : le Parlement doit pouvoir exercer

Nous accueillons avec bienveillance les modifications apportées au cadre pluriannuel des finances publiques, en particulier la fixation d'une norme pluriannuelle de dépenses des administrations au sein des lois de programmation. Pour autant, ce nouveau cadre que constitue la pluriannualité ne satisfait pas encore entièrement à la démarche de performance et à la logique de résultat qui irriguent la LOLF. Les lois de programmation pourront toujours être remises en cause chaque année, la proposition sénatoriale visant à permettre l'adoption de lois de programmation des finances publiques rectificatives en cas d'objectifs macroéconomiques caducs n'ayant pas été retenue. Concernant l'ajustement du calendrier budgétaire, ce texte prévoit la mutualisation du débat sur le programme de stabilité et du débat sur le rapport d'orientation des finances publiques pour permettre un « printemps de l'évaluation ». Cette continuité renforcée du chaînage budgétaire est à saluer. Dans cette même optique, la proposition de loi organique prévoit la création d'une nouvelle catégorie de loi de finances : la loi de finances de fin de gestion. Elle remplacera la loi de finances rectificative, désormais habituelle en fin d'exercice, sans permettre l'inscription de mesures fiscales nouvelles.

L'insertion dans nos textes budgétaires de trois scénarios d'évolution des taux d'intérêt mesurant leur impact respectif sur la charge de la dette est à souligner. Nous ne pouvons toutefois que regretter que l'amendement visant à instaurer une annexe spécifique récapitulant, sous forme de tableaux, le nombre de postes rémunérés par l'État au moment du débat budgétaire et leur variation pluriannuelle n'ait pas été retenu les instruments actuels ne permettent pas d'obtenir une vue générale et synthétique, consignée dans un même document, pour l'ensemble des missions budgétaires et par ministère. Enfin, ce texte améliore la procédure d'examen du budget en prévoyant notamment que l'ensemble des recettes soient appréciées en première partie. La Haute Assemblée a également adopté une mesure tendant à plafonner les reports de crédits, hors cas de nécessité impérieuse d'intérêt national, et à renforcer les exigences de motivation applicables à ces dérogations afin de préserver le principe cardinal d'annualité. Le groupe Union Centriste souscrit à ces évolutions substantielles de la LOLF, qui s'appliqueront à l'examen du projet de loi de finances pour 2023. Elles laissent espérer que l'après-crise ne fasse pas du « quoi qu'il en coûte » la règle pour les comptes publics.

À cet égard, je ne peux que renouveler les regrets que le président Requier a émis hier, au nom de notre groupe, après le rejet par la majorité sénatoriale de la première partie du projet de loi de finances pour 2022. de finances pour 2022. L'issue conclusive de ces commissions mixtes paritaires est bienvenue, vingt ans après l'adoption de la LOLF. Elle prouve la capacité de nos deux assemblées à travailler de concert pour améliorer la visibilité de nos finances publiques. publiques. Je tiens à remercier les présidents de chacune des commissions des finances de nos deux assemblées, ainsi que les rapporteurs généraux, sans qui nous n'aurions pu aboutir à ces textes d'équilibre. Probablement pourrons-nous tous nous accorder sur l'objectif annoncé : redonner du sens à la programmation pluriannuelle de nos finances publiques

Cette lisibilité, nous la devons à l'ensemble de nos concitoyens, en vertu de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dispose que « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique [

est du contenu, nous sommes favorables à la fixation d'une norme pluriannuelle de dépenses des administrations publiques. Le respect du calendrier des deux assemblées dans l'organisation des différents débats de nature budgétaire- sur le programme de stabilité, sur l'orientation des finances publiques,

Mon groupe, attaché au débat et aux droits des parlementaires, ne peut que regretter les limites qu'oppose l'article 40 de la Constitution à notre droit d'amendement. Les irrecevabilités nous ont enfermés dans un simple pouvoir d'alerte en matière budgétaire ; nous ne pouvons nous y résoudre.

du Gouvernement, l'ensemble de la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.